la gestion des crises de manière générale, au-delà de cet enjeu de court terme ; la hausse des prix de l'énergie, qui demeure une préoccupation centrale en Europe

Face à cette cinquième vague, nos priorités sont bien identifiées et, je crois pouvoir le dire, la coordination européenne, forte des leçons tirées des précédentes vagues de covid-19, s'est améliorée.

mois : six mois après la vaccination complète, avec trois mois de marge accordée aux États membres pour imposer ou non une plus ou moins grande restriction d'accès. Il importe, ensuite, de renforcer la couverture vaccinale, en ciblant les personnes qui n'ont pas encore été vaccinées et en généralisant, comme nous le faisons partout en Europe, avec un approvisionnement significatif, les doses de rappel. Enfin,

des affaires étrangères du Sénat, Christian Cambon, s'est d'ailleurs rendue récemment en Pologne afin d'échanger notamment sur les sujets et les enjeux de sécurité et de défense dans la perspective de la présidence française de l'Union européenne ; je veux saluer ces travaux du Sénat.

Nous avons aussi, nous le savons, nos propres difficultés. Nous avons vécu nos propres drames, comme celui qui a coûté la vie à vingt-sept personnes voilà quelques jours Cela montre aussi que sur ce sujet une coopération européenne est indispensable pour partager le renseignement et démanteler les filières de passeurs. Tel fut l'objet de la réunion organisée par le ministre de l'intérieur à Calais juste après ce nouveau drame.

Je l'ai dit, nous avons réussi à mener une action commune qui a contribué à la désescalade. J'évoquais aussi le dialogue avec les pays tiers, notamment la Russie

Conseil européen : celle de l'Éthiopie. Alors que la situation sur le terrain continue d'évoluer de manière préoccupante et sans qu'un camp prenne le dessus sur l'autre par les armes, nous continuerons d'appuyer tous les efforts engagés pour parvenir à un cessez-le-feu.

17 décembre prochains sera, sauf événement très exceptionnel, la dernière avant le début de la présidence française. À cet égard, nous avons une responsabilité particulière, de préparer dans les meilleures conditions possible la mise en oeuvre de nos priorités, qui sont nombreuses, au cours du premier semestre de l'année prochaine. Dans ce contexte, j'aimerais attirer votre attention sur trois enjeux qui seront évoqués lors de cette réunion réunion et dont la commission des affaires étrangères et de la défense assure un suivi particulièrement actif. En premier lieu, pour ce qui concerne notre dialogue avec le Royaume-Uni, il est temps, monsieur le secrétaire d'État, que les Britanniques tiennent parole et mettent en application les termes de l'accord de commerce et de coopération conclu le 24 décembre 2020. Il s'agit non seulement d'une question de confiance entre nous et le Royaume-Uni, mais également d'une question de crédibilité pour les institutions de l'Union : celles-ci ne sauraient détourner le regard face un partenaire qui ne cesse, depuis plusieurs mois, de remettre en cause verbalement et matériellement les engagements souscrits dans le cadre de cet accord. En ce qui concerne l'Irlande du Nord, cela fait maintenant plus d'un mois que la Commission a rendu publiques ses propositions d'aménagement à l'application du protocole nord-irlandais. J'espère que vous serez en mesure de nous expliquer quel est l'état actuel des négociations et quelle voie de sortie est envisageable, s'agissant d'un partenaire qui n'a pas abandonné sa menace régulièrement réitérée

Parallèlement, monsieur le secrétaire d'État, nous attendons de vous des réponses claires et un calendrier précis quant à la mise en oeuvre déjà maintes fois repoussée des stipulations de cet accord en matière de pêche. Nous savons bien que le Président de la République a fixé comme délai limite la date du 10 décembre pour faire aboutir ces négociations, mais, à quarante-huit heures de cette date et après plusieurs mois de négociation, nous espérons que vous serez en mesure de dresser pour nous un état des lieux circonstancié des avancées que vous avez obtenues

qui pèsent sur les frontières de l'espace Schengen. À cet égard, nous attendons des précisions sur la position de la France dans le débat que la Commission et le haut représentant Borrell ont ouvert, le 23 novembre dernier, en présentant une communication sur la réponse à apporter à l'instrumentalisation par des États des mouvements migratoires aux frontières de l'Union. En particulier, monsieur le secrétaire d'État, si nous ne pouvons que nous réjouir de la stabilisation progressive de la situation à la frontière biélorusse, comment ferons-nous pour empêcher qu'une nouvelle attaque hybride de ce type ne se reproduise à nos portes ? Il est essentiel que vous puissiez nous apporter des précisions sur la position française dans le cadre de la réforme à venir du code frontières Schengen.

En vue de la présentation d'une nouvelle version de ce document le mois prochain, quels amendements le Gouvernement entend-il y apporter ? Plus précisément, quelle articulation la France propose-t-elle entre la garantie apportée par l'OTAN et l'autonomie stratégique de l'Union,

par des fonds européens ? À quelques semaines du début de la présidence française du Conseil de l'Union, les enjeux- vous l'avez dit -sont nombreux. Ce dernier sommet de l'année 2021 doit nous permettre de prendre clairement position et nous mettre en situation d'assumer pleinement nos priorités stratégiques

ainsi que sur les prix de l'énergie, deux sujets que suit avec attention la commission des finances. Alors que les promesses d'une reprise économique vigoureuse étaient en passe d'être concrétisées, l'OCDE,

de vue économique, le plan de relance européen représente un soutien incontestable. J'ai bien noté que la transition énergétique a été définie comme une orientation forte, conformément au Pacte vert pour L'on peut s'en réjouir, mais il ne faudrait pas que la réglementation européenne sur la « taxonomie », c'est-à-dire la classification des activités économiques selon leurs effets sur l'environnement définie par le règlement européen adopté en 2020, vienne à pénaliser la France en classant le nucléaire parmi les activités ne relevant pas de la catégorie dite durable. Absolument ! Les atouts économiques, technologiques et environnementaux dont nous disposons dans ce domaine ne doivent pas être sacrifiés sur l'autel de l'idéologie ou d'un consensus mou. Pouvez-vous nous rassurer sur ce point ? La flambée du coût de l'énergie pose le problème du pouvoir d'achat des ménages. Les dispositions prises par le Gouvernement étant conjoncturelles, elles ne sauraient constituer une réponse dans la durée. Ainsi le « bouclier tarifaire » destiné à contenir les prix du gaz et de l'électricité apparaît-il d'ores et déjà insuffisant. Le dispositif prévu pour limiter à 4 % la hausse des prix de l'électricité coûtera beaucoup plus cher que prévu et risque fort de ne pas suffire. Des experts estiment que son coût budgétaire pourrait dépasser 10 milliards d'euros quand le rendement total de la taxe sur l'électricité, qu'il est d'ailleurs prévu de minorer, est inférieur à 8 milliards d'euros La hausse sans précédent des prix de l'énergie n'est pas sans lien avec le marché européen de l'énergie, ainsi qu'avec le système d'échange de quotas d'émission de l'Union. En effet, l'augmentation du prix de l'électricité résulte directement de la hausse du prix du gaz, les prix de ces deux énergies étant liés au sein dudit marché européen de l'énergie.

quelques divergences apparues au sein du Gouvernement, la France a pris l'initiative d'une proposition de réforme d'ampleur du marché européen de l'électricité. Si quelques pays s'y sont ralliés- je pense à l'Espagne, à l'Italie, à la Grèce et à la Roumanie

alors que les divergences entre les Vingt-Sept promettent d'être à nouveau très prononcées sur le sujet de la réforme du marché de l'électricité, comment la France entend-elle promouvoir ce projet dans les mois à venir, en particulier dans la perspective de sa prochaine présidence du Conseil ?

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, je vous prie tout d'abord d'excuser le président de la commission des affaires européennes, Jean-François Rapin qui, en déplacement en Grèce avec le président du Sénat, m'a chargé de le représenter ce soir. La prochaine réunion du Conseil européen sera la première pour le nouveau chancelier allemand, intronisé aujourd'hui même par le Bundestag. C'est une bonne nouvelle pour l'Union européenne que l'Allemagne soit parvenue, en moins de deux mois, à se doter d'une coalition et que celle-ci se soit accordée sur un programme converge avec les priorités que nous espérons précisément voir prospérer sous la présidence française du Conseil, à compter du 1 janvier 2022 : « accroître la souveraineté stratégique de l'Union européenne » et mieux défendre les « intérêts européens communs précieux motif d'espoir, vu le contexte par ailleurs assez sombre dans lequel se déroulera la réunion du Conseil européen dans huit jours. De nouveau, le sujet de la pandémie de covid-19 revient à l'ordre du jour et, avec lui, l'impératif d'une coordination des mesures aux frontières intérieures et extérieures de l'Union, après l'activation du frein d'urgence qui a consisté à suspendre les vols en provenance d'Afrique australe. La question se pose de savoir comment préserver la liberté de circulation, compte tenu de la disparité de la couverture vaccinale entre États membres. Monsieur le secrétaire d'État, pouvez-vous nous dire si le Conseil européen abordera l'hypothèse de l'obligation vaccinale, qui émerge dans plusieurs États

Il est essentiel de trouver le moyen d'améliorer les mécanismes du marché de détail de l'électricité, afin de stabiliser les prix et d'inciter à la consommation d'énergie bas-carbone. Cette réunion n'y suffira sans doute pas, mais le cas d'Ascoval, qui a failli délocaliser en Allemagne sa production d'acier pour bénéficier d'une électricité moins chère, mais bien plus polluante, montre qu'il y a urgence à relever ce défi.

de l'énergie nucléaire dans cette taxonomie, car il s'agit d'une énergie bas-carbone, mais également abondante, peu chère et régulière. L'enjeu est de permettre à l'Union européenne d'atteindre la neutralité carbone en 2050 et de conforter son autonomie stratégique,

de décembre sera donc l'occasion d'un premier échange permettant d'évaluer dans quelle mesure les États membres partagent la même vision des menaces et la même ambition pour y répondre ensemble.

assez ambivalent, puisqu'il sera à la fois celui de la campagne électorale, ce qui ne saurait échapper à personne, et celui de notre présidence du Conseil de l'Union, dont il serait bon qu'elle soit marquante. D'autre part, nous subissons toujours les vagues pandémiques ; les variants mettent au jour nos fragilités sanitaires, sociales et économiques. En outre, nous voyons malmenées à nos frontières et sur nos côtes les valeurs qui ont fondé le projet européen. Sur le front climatique, la COP26, les accords commerciaux, la politique agricole commune (PAC) ou la question de la taxonomie pour une finance durable montrent combien les politiques écologiques sont à la peine face aux dénis, aux atermoiements et aux lobbies à courte vue. moment est aussi celui où une nouvelle coalition allemande pose les bases d'une nouvelle donne. N'est-ce pas là une forte raison de plus pour redonner vigueur au projet européen commun ? Face au covid-19, l'Europe est d'autant plus attendue qu'elle est par nature vouée à la coopération et à la solidarité, en interne, mais aussi au niveau international, où se joue, on le sait, l'essentiel. On pourrait certes se borner à ressasser que l'Europe a su mutualiser sa production et sa distribution vaccinales, qu'elle fournit beaucoup de doses aux pays pauvres et qu'en comparaison avec les autres privilégiés nous ne sommes pas les plus égoïstes, mais ces satisfecit même justifiés, ne changeront pas la donne sanitaire planétaire : seule une infime part des près de 6 milliards de doses injectées dans le monde est allée à des pays à faibles revenus. Face aux drames humains et aux fabriques à variants, si l'on veut réduire les coûts et porter la production vaccinale à la hauteur des besoins planétaires, la levée des brevets et les transferts de savoir-faire et de technologies sont impératifs. En la matière, l'Europe est- je le répète -d'autant plus attendue qu'elle n'est pas la moins bonne parmi les acteurs décisifs. Redonner vigueur au projet européen passera également par une réforme profonde de notre politique migratoire, qui met en difficulté, et c'est un euphémisme, tant les pays d'entrée que, surtout, les personnes exilées. Le tout-sécuritaire et la sous-traitance à des États tiers de la tenue des frontières par les armes défont la dignité humaine et les valeurs qui nous constituent. Sortons de cette logique de protection des frontières qui ne protège pas les droits des personnes, déployons des moyens humanitaires partout où la vie humaine est menacée, ouvrons des voies de migration sûres et légales, instaurons un mécanisme efficace de relocalisation et de solidarité financière entre les États afin de faciliter l'accueil, l'intégration et le traitement de l'asile conformément aux exigences du droit international. Autre sujet : la directive sur le salaire minimum met en jeu les droits sociaux, et en particulier le droit à un revenu décent.

Soyons clairs : la question des déchets radioactifs et des risques majeurs empêche l'activité nucléaire de satisfaire aux critères de la durabilité ; il ne s'agit pas d'idéologie, mais de cohérence ! Et si un « » incluant le gaz fossile devait éviter le possible rejet par une majorité qualifiée,

qu'il faut ménager à l'industrie automobile pour éviter le désastre social. Concluant ce rapide exposé de nos préoccupations et propositions principales à la veille de cette réunion du Conseil européen, j'ajouterai que, pour renforcer la position internationale de faire passer le commerce international du libre-échange au juste échange. La politique commerciale de l'Union comme outil de régulation au service du climat et de la transition écologique, voilà la voie à consolider.

La politique migratoire de l'Europe est un naufrage, indigne des enjeux de sécurité humaine globale qui sont ceux de notre époque. Ces dernières semaines, l'instrumentalisation inacceptable par la Biélorussie de quelques milliers de migrants est devenue l'arbre qui cache la forêt de cette indignité européenne. Ces migrants seraient donc, selon la terminologie vulgarisée par les dirigeants polonais et européens, une « arme » au service d'une « guerre hybride » visant la déstabilisation de l'Union. Soyons sérieux ce chantage, comme ceux de la Turquie, du Maroc, du Royaume-Uni et d'autres, n'a de poids que parce que l'Union européenne referme partout ses portes aux voies légales et sécurisées de migration, poussant à la concentration de migrants aux frontières, livrant ceux-ci aux marchandages des passeurs. Les enjeux humains et politiques ont laissé place à un lexique militaire et sécuritaire qui enfonce l'Europe dans le déni des défis humains du XXI siècle. Un rapport de l'institut Jacques-Delors publié voilà quelques jours fustige d'ailleurs « un conflit profond de valeurs qui tend à opposer le besoin de sécurité des citoyens européens aux idéaux sur lesquels se fonde leur appartenance à l'Union européenne. La politique d'accueil et le droit d'asile sont maltraités comme jamais par les pays membres de l'Union européenne. Nous ne traitons sérieusement aucune des causes profondes des migrations forcées : ni les guerres, auxquelles nous participons activement,

ni les écarts grandissants de richesses, dont le Laboratoire des inégalités mondiales vient de dresser un tableau alarmant ; ni les grands trafics criminels. Nous n'abordons pas plus ambitieusement les enjeux vertueux d'une circulation des personnes, des jeunes, des savoirs, des cultures. Or qu'est-ce qui est le plus digne et le plus fécond pour l'avenir ? Accueillir plusieurs milliers de migrants afghans après le fiasco du départ américain de Kaboul, comme nous venons de le faire et comme nous devons continuer de le faire, ou bloquer ces Afghans aux frontières en les livrant aux passeurs et aux démagogues ? Oui, les voies sécurisées de migrations sont plus sûres pour tous, pour les migrants comme pour les Européens. Ce n'est pas le déferlement qui nous menace, ce sont l'égoïsme, la peur et le repli.

Ceux-là mêmes qui ont défendu la libéralisation et la globalisation en viennent à crier au loup sur les interdépendances, c'est un comble ! Selon les auteurs de cette boussole stratégique, tout est conflictualité et l'OTAN et sa logique de confrontation permanente semblent constituer un horizon indépassable.

trancher enfin en faveur de la levée des brevets. Cette solution s'impose à un point tel que le Parlement européen a adopté une résolution réclamant la levée temporaire des brevets sur les vaccins le 25 novembre dernier. La Commission européenne et les États membres récalcitrants campent sur le principe

ce temps, les laboratoires Pfizer, BioNTech et Moderna annoncent un bénéfice annuel avant impôts de 34 milliards d'euros, correspondant à un profit combiné de 65 000 dollars par minute. Il faut taxer les Big Pharma

La France pourrait soutenir cette proposition. Enfin, de manière plus large, en Europe même, les règles et les critères de financement pour la relance d'une nouvelle vision économique doivent être bouleversés. (BCE) doit libérer les États de la charge des 20 % de titres de dette publique qui sont désormais en sa possession et le pacte de stabilité doit être abandonné au profit d'un pacte de financement social et écologique.

personnes qui se lancent, à leurs risques et périls, dans une dangereuse traversée, avec l'espoir d'une vie meilleure. Nous devons les protéger des passeurs, qui exploitent cette détresse.

Tous les États doivent donc prendre leurs responsabilités. Si la France est en première ligne sur cette question, car les départs s'effectuent depuis nos côtes, il est impératif que tous les États membres s'impliquent, notamment pour contenir plus efficacement plus efficacement les mouvements secondaires au sein de l'espace Schengen. La semaine dernière, nous avons appris que le Royaume-Uni avait signé une déclaration conjointe visant à renforcer la coopération avec la Belgique, en particulier dans le cadre de la lutte contre l'immigration illégale.

des mesures doivent être adoptées pour améliorer le cadre juridique de protection contre l'exploitation et des sanctions contre les passeurs, et pour mettre en place des partenariats opérationnels. Monsieur le secrétaire d'État, pourriez-vous nous préciser l'avancée du processus d'adoption de ces mesures et de la révision des règlements existants ?

Ce type d'accord prévoit une coopération avec l'État d'origine pour que les personnes y soient réadmises. Un tel accord avec le Royaume-Uni aurait pour but de faciliter le retour en France des personnes entrant sur le territoire britannique depuis le territoire français.

Dans quelle mesure nos partenaires européens sont-ils mobilisés sur cette question, notamment à la suite de la réunion qui s'est tenue à Calais ? Je conclurai un dernier point d'interrogation, tant les questions sont nombreuses depuis le Brexit, relatif à la politique de défense. En quittant l'Union européenne, le Royaume-Uni est sorti de la politique de sécurité et de défense commune et l'accord de commerce l'accord de commerce et de coopération, signé l'année dernière, ne mentionne pas ce volet. Or le Royaume-Uni reste un membre important et actif de l'OTAN.

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, la question des migrations est revenue de façon brutale sur le devant la scène européenne en raison du naufrage d'une embarcation, non loin de nos côtes, qui a causé la noyade dramatique de 27 migrants.

il est dans l'intérêt de tous les États membres de coopérer et de mobiliser les moyens opérationnels adéquats. Il convient en outre de ne pas oublier les valeurs fondatrices de l'Union européenne, au premier rang desquelles figure la solidarité.

situation, la prévention demeure fondamentale. À cet égard, l'Europe doit envoyer un message politique ferme à tous ceux qui facilitent directement ou indirectement les migrations. Je pense d'abord et surtout à l'instrumentalisation des migrants comme arme de pression politique. de sa réunion des 21 et 22 octobre derniers, a condamné les attaques hybrides menées aux frontières de l'Union européenne et a déclaré vouloir y réagir en conséquence. Comment la France s'emparera-t-elle de ce sujet lors de sa prochaine présidence ? Où en sont les huit plans d'action pour les pays d'origine et de transit promis par la Commission européenne voilà quelques mois ? Enfin, si tout doit être mis en oeuvre pour éviter les drames humanitaires, l'Europe doit

Le projet de règlement du Conseil pour une gestion commune des contre-mesures médicales en cas de crise sanitaire transfrontalière est en route et c'est une bonne chose.

veux souligner l'intérêt que nous aurions au fait de garantir le plus rapidement possible la souveraineté européenne en matière de production de médicaments. Notre dépendance à l'égard de pays tiers pour la production de principes actifs et de certains équipements médicaux doit être rapidement réduite.

l'occasion pour souligner que ces tensions sur l'énergie pourraient s'aggraver si les États membres n'arrivaient pas à s'accorder sur les orientations de la taxonomie. La résolution européenne sur l'inclusion du nucléaire dans le règlement délégué

Il s'agit à la fois de contribuer à décarboner les sources d'énergie à long terme, mais aussi de limiter la flambée des prix qui nous préoccupe actuellement. En marge de l'agenda de la prochaine réunion du Conseil européen, je veux évoquer une dernière question, qui n'est pas sans lien avec la précédente. En ce qui concerne les conséquences de la pandémie de covid-19 sur l'économie, la situation est très contrastée et évolue

belgo-espagnole d'un mécanisme d'alerte en cas de déséquilibre social, à l'instar de ce qui existe pour les déséquilibres macroéconomiques. L'Union européenne doit en effet promouvoir des exigences fortes en matière de politique sociale et d'emploi. Dans cette perspective, il faut veiller à ce que les bénéfices de la relance soient équitablement partagés. Sans cela, faute de solidarité et de convergence, l'Europe échouera à construire un projet véritablement inclusif et vecteur d'espoir pour tous nos concitoyens.

C'est dans les épreuves que l'on mesure la solidité des organisations. Force est de le constater, ce ne sont pas les crises qui manquent et de fortes turbulences ne cessent de mettre à l'épreuve nos institutions. Les élus littoraux, dont je fais partie, savent bien que la conjonction des vents et des marées est propice à l'érosion du trait de côte et aux catastrophes engendrées par les submersions marines. Face à ces menaces, trois stratégies sont possibles : le renforcement de nos défenses, l'adaptation ou le repli. Le résultat du référendum britannique du 23 juin 2016 a fait l'effet d'un tsunami, dont on pouvait estimer les conséquences et s'y préparer : en effet, la procédure prévue à l'article 50 du traité sur l'Union européenne offrait du temps, avant que la vague n'arrive sur nos côtes, pour négocier et conclure un accord de retrait ainsi qu'un accord commercial et de coopération.

Ainsi, les Britanniques ont acquis implicitement la maîtrise du calendrier, imposant, à coups de psychodrames, leur propre tempo, jusqu'à aboutir, de report en report, à un accord de dernière minute, conclu fin décembre 2020, qui comportait de nombreuses zones d'ombre. Le cas des licences de pêche est très emblématique. En la matière, l'accord n'est pas respecté. En février dernier, le Royaume-Uni a fixé, de façon unilatérale, de nouvelles conditions d'éligibilité notamment la preuve de l'antériorité au moyen de données de géolocalisation. Il a en outre imposé des conditions sur les espèces, sur les jours de pêche et sur les techniques utilisées, afin de restreindre l'activité de ceux qui avaient obtenu des licences. Depuis plus de dix mois,

les négociations s'enlisent et les sanctions annoncées à grand renfort de rodomontades ont été différées par le Président de la République en marge de la COP26, selon le principe suivant lequel ce n'est pas pendant que l'on négocie que l'on va infliger des sanctions, oubliant que les Britanniques ont inventé la négociation perpétuelle et le Brexit sans fin ... L'erreur de communication de la ministre de la mer sur les mesures compensatoires et l'activation

Monsieur le secrétaire d'État, alors que les droits historiques et les droits issus de l'accord de retrait sont bafoués, quelle réaction forte proposez-vous d'inscrire à l'agenda européen ? À quel moment et selon quelles modalités faudra-t-il activer l'instance de règlement des différends de l'accord post-Brexit ?

ait lieu, l'horreur de la mort par noyade de 27 migrants à laquelle s'est ajoutée une nouvelle provocation de Boris Johnson, qui proposait le retour sur le sol européen des migrants en situation irrégulière.

pour lutter efficacement contre les passeurs et contraindre la Grande-Bretagne à ouvrir davantage les voies de migration légale ? À la frontière biélorusse, ce sont les valeurs de l'Union européenne qui sont mises en péril. La première nécessité est de venir en aide à ceux qui ont été instrumentalisés par le régime biélorusse et qui sont aujourd'hui piégés. De même, l'utilisation d'êtres humains comme arme de guerre hybride et asymétrique doit être condamnée et les instigateurs durement sanctionnés devant une cour internationale. Les opérateurs de transport qui se sont rendus complices ou ont manqué de vigilance face à de telles pratiques doivent également faire l'objet de mesures spécifiques. L'attitude la Pologne ne laisse pas non plus de susciter des interrogations. La solution ne passe ni par un refoulement systématique ni par l'édification d'un mur infranchissable. L'accès aux abords de la frontière biélorusse doit être garanti aux journalistes et aux associations humanitaires, qui ont respectivement pour missions d'informer d'informer et de secourir. La menace de saisine de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) et le déploiement d'une structure d'enregistrement des demandes d'asile seraient de nature à inciter la Pologne à respecter ses obligations en la matière. Enfin, il semble inopportun il semble inopportun que de l'argent européen puisse être mobilisé pour financer un mur de protection, symbole d'un repli frileux. En évoquant le plan de relance européen, Thierry Breton disait que « l'Europe avance avec des crises ». Souhaitons

J'ai appris hier que l'Assemblée nationale organiserait un débat sur ce sujet la semaine prochaine, mais j'ai cru comprendre que ce ne serait pas le cas à la Haute Assemblée.

j'ai eu deux longs entretiens avec des eurodéputés allemands, qui, connaissant sans doute mal le fonctionnement politico-institutionnel de notre pays, s'imaginaient que j'étais en mesure de leur apporter quelque éclairage.

éventuelles déceptions liées à des attentes disproportionnées au regard de ce qu'est réellement, aujourd'hui, la présidence tournante du Conseil européen.

permanente du Conseil européen, la présidence française sera également largement encadrée par le système du trio de présidences, supposé assurer une continuité entre trois présidences tournantes successives.

La présidence qui vient devra en premier lieu faciliter l'adoption définitive d'un certain nombre de textes déjà programmés et en faire avancer d'autres, sur des sujets encore très discutés, tels que la directive relative au devoir de vigilance

pour définir de nouvelles lignes directrices, non pas seulement à l'horizon de ses six mois de mandat, mais bel et bien pour les dix-huit mois à venir. Elle aura, à ce titre, plus que son mot à dire sur les chantiers à engager et à poursuivre lors des présidences tchèque et suédoise, qui suivront.

d'un alignement favorable des planètes, au sein de la « constellation Europe », il était bon d'avoir connaissance du contrat de coalition négocié par nos amis allemands. Or c'est chose faite depuis la fin du mois de novembre et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce texte de 177 pages, contraignant pour ses parties signataires, met en lumière bien des convergences de vue entre nos deux pays sur les défis européens d'aujourd'hui et de demain,

C'est là un excellent présage, non seulement pour la prochaine présidence française, mais surtout pour les quatre années à venir. Comme j'entends rester optimiste quant à l'avenir de l'Europe, je vois aussi un autre présage positif dans l'annonce, le 1 décembre dernier, par la présidente de la Commission, du projet, consistant en un financement, financement, à hauteur de 300 milliards d'euros, d'infrastructures durables dans les Balkans et en Afrique, pour contrer les nouvelles routes de la soie lancées voilà plus de huit ans par la Chine.

par « passerelle mondiale ». Après les autoroutes de l'information des années 1990 et les routes de la soie des années 2010, on pourrait ironiser en disant que, avec sa « passerelle », l'Union européenne des années 2020 entre dans l'ère dans mobilités douces ... On peut aussi s'interroger sur la pertinence du montant prévu et sur la faisabilité d'un tel projet au regard des exigences posées en matière de gouvernance, de transparence, de respect des valeurs démocratiques, de partenariats équitables et d'objectifs de neutralité climatique et de développement durable, mais ne faisons pas la fine bouche : c'est une initiative, certes mais qui prend enfin en compte la nouvelle donne géopolitique mondiale. Compte tenu du moment où elle a été annoncée, j'imagine que la Commission européenne a dû consulter en amont les autorités françaises et la nouvelle majorité allemande. Monsieur le secrétaire d'État, vous qui en savez certainement plus que nous à ce sujet,

monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, lors d'un énième tour de négociation, Donald Tusk, ancien président du Conseil européen, alertait sur la nature même du Brexit, en déclarant que « le plus dur, ce n'est pas la séparation, c'est la construction d'une nouvelle relation après la séparation. » Or c'est bien une étape cruciale de cette nouvelle relation que nous vivons actuellement de part et d'autre de la Manche et, autant le dire, pour le moment, elle ne prend pas le bon chemin Depuis le début de l'application de l'accord du Brexit, on ne peut d'ailleurs pas dire que les Britanniques jouent franc-jeu, ce qui fait craindre bien des complications à moyen et long termes. Nous devons, nous Européens, rester fermes et solidaires. Je dis « solidaires », car, parfois, l'Union européenne manque de voix. Sur le dossier des licences de pêche par exemple, le groupe Les Indépendants a appelé, lors de la séance des questions d'actualité au Gouvernement du 24 novembre dernier, à un engagement fort de la Commission européenne.

récents et tragiques événements, un autre dossier requiert la concertation et l'intervention de l'Union européenne : la crise des migrants dans la Manche. Nous devons trouver des solutions à cette situation urgente, qui a déjà coûté la vie à trop de personnes,

Je salue cette volonté de travailler ensemble contre les passeurs et leurs filières : ces personnes mettent en danger la vie des gens pour de l'argent et c'est inacceptable ! Il faut que ce dossier soit plus « européanisé », puisqu'il concerne, même indirectement, Monsieur le secrétaire d'État, envisagez-vous d'aborder ce sujet lors du Conseil européen ? Le pacte européen sur la migration et l'asile est-il une priorité de la présidence française de l'Union européenne ?

La Commission avait mis en place une boîte à outils, dont l'objectif était de contrer cette augmentation rapide des tarifs et de permettre aux États de réagir vite, mais cette réponse est de très court terme et les intérêts des pays européens sont assez divergents, particulièrement en ce qui concerne la révision du marché intérieur

La cinquième vague a submergé les États membres de l'Union européenne, où les courbes de contaminations montent en flèche. Alors que, dans de nombreux pays, la vaccination est le sujet majeur, où en sommes-nous des négociations autour de la construction d'une Union de la santé ?

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, à l'occasion de la prochaine réunion du Conseil européen, les chefs d'État et de gouvernement se pencheront sur la préparation du sixième sommet entre l'Union européenne et l'Union africaine. Il s'agira d'un rendez-vous important, notamment pour progresser sur la voie d'un partenariat économique renouvelé, à la fois plus robuste et plus équilibré. En effet, un changement de paradigme est désormais nécessaire pour dépasser la seule logique de l'aide au développement et favoriser les investissements, en particulier dans les compétences, la croissance des entreprises et, plus largement, la transformation déjà amorcée des économies africaines. Ce sommet sera également l'occasion d'aborder la crise sanitaire. En tant que président du groupe sénatorial d'amitié France-Afrique de l'Ouest, j'ai pu constater, lors d'un récent déplacement au Bénin et au Togo, que, si l'Afrique demeure relativement épargnée par rapport à d'autres régions du monde, la covid-19 y a néanmoins des répercussions fortes, qui font peser de nombreuses incertitudes sur sa stabilité et sa prospérité. Or, pas plus en Afrique qu'en Europe, il n'existe de solution miracle et la vaccination massive demeure le moyen le plus sûr de vaincre le virus. Dans cette optique, la Commission européenne et les États membres se sont mobilisés pour conforter la réponse africaine à la crise. Un nouvel appui financier d'au moins 1 milliard d'euros a ainsi été annoncé au mois de mai dernier pour soutenir le développement des capacités sanitaires africaines, la fabrication locale de vaccins et la planification logistique des campagnes de déploiement. Par ailleurs, dans le cadre de l'initiative Covax, 700 millions de vaccins ont été promis d'ici au milieu de l'année prochaine

Réduire cette fracture vaccinale croissante est une obligation morale, mais ne perdons pas de vue que cette solidarité va aussi dans le sens de notre propre intérêt, puisque nous voyons bien, avec le variant omicron, qui est apparu en Afrique du Sud et qui gagne désormais nos latitudes, que, tant que l'humanité entière ne sera pas aussi bien protégée que possible, notre continent demeurera lui aussi vulnérable. Autre sujet pour lequel une coopération euro-africaine plus étroite et plus efficace est incontournable : la gestion des flux migratoires,

Je souhaite insister sur cet aspect, car la mise en oeuvre de retours efficaces est une composante fondamentale de la crédibilité d'une politique migratoire européenne, qui a par ailleurs toutes les peines du monde à voir le jour. Or les résultats en la matière, sévèrement épinglés par la Cour des comptes européenne, sont- il faut le dire -catastrophiques. À peine 29 % des personnes qui se voient délivrer chaque année l'ordre de quitter le territoire de l'Union regagnent effectivement leur pays ; cette proportion tombe même à 19 % si l'on exclut du calcul les ressortissants des Balkans occidentaux. Le signal envoyé est délétère Une fermeté accrue dans notre dialogue avec les pays d'origine est donc indispensable. Cela étant, dans ce contexte, une voie encore peu empruntée mériterait de l'être davantage celle des retours volontaires. En effet, les retours sont plus efficaces et moins coûteux quand ils peuvent se dérouler sur une base volontaire et s'accompagner de véritables chances de réintégration.

qui charge notamment Frontex d'assister les États membres dans le développement de l'aide au retour volontaire, est une bonne base de départ. Toutefois, si les initiatives envisagées vont dans le bon sens, le programme européen reste flou concernant la prise en charge financière de l'aide au retour et, surtout, les incitations concrètes, financières ou non, qui pourraient encourager les pays d'origine à s'engager véritablement dans un processus de réadmission et de réintégration. Plusieurs options sont actuellement étudiées, mais il faudra, en tout état de cause, avancer avec nos partenaires africains sur ce dossier, si nous voulons une politique européenne de retour enfin efficace et durable. Pour conclure, je souhaite aborder un dernier axe majeur du prochain sommet Europe-Afrique, à savoir l'indispensable coopération sécuritaire, notamment dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Avec les opérations Serval puis Barkhane, la France est en première ligne de ce combat depuis maintenant près de neuf ans. Elle est en première ligne, mais surtout bien seule et, de surcroît, en butte à une défiance croissante des populations locales, parfois instrumentalisées par tous ceux qui ont un intérêt à l'effacement de la France dans cette région. Tout charge de la lutte contre les groupes djihadistes par les pays de la bande sahélo-saharienne reste, malgré les efforts de ces pays et la formation du G5 Sahel, bien en deçà de ce qui serait nécessaire.

Avec la refonte du dispositif militaire français, la est appelée à tenir un rôle plus important. Il est indispensable que cette montée en puissance se confirme et que davantage de pays européens y contribuent à la fois en hommes et en matériel. La parole est à Mme Catherine

-de trouver des solutions permettant de résoudre les graves dysfonctionnements qui les caractérisent désormais. En réalité, elles ont même démontré tout le contraire, comme l'ont bien mis en évidence les révélations de la lanceuse d'alerte Frances Haugen, que nous avons entendue en audition au Sénat, le 10 novembre dernier.

et l'évaluation de tous les types de risques, selon des protocoles établis par les chercheurs et les régulateurs, et non par les plateformes elles-mêmes. Ces dernières ne devraient pas non plus pouvoir opposer le secret des affaires aux autorités de régulation et aux chercheurs agréés par ces autorités. En effet, qu'étant des acteurs privés, ces grandes plateformes sont devenues des quasi-infrastructures publiques, ce qui justifierait de nouveaux modes de régulation, adaptés aux caractéristiques propres à l'espace en ligne. L'espace en ligne n'est pas identique à l'espace public dans le monde réel, car il est déformé par l'amplification algorithmique. La lutte contre les propos illicites devrait donc s'accompagner de mesures visant à lutter spécifiquement contre leur viralité. En d'autres termes, il faut encadrer les modalités de diffusion, le « », comme disent les plutôt que les contenus eux-mêmes, le « ». Surtout, ne nous laissons pas enfermer dans le piège qui consiste à dire qu'il faut s'attaquer aux contenus, et ce au détriment de la liberté d'expression. En sélectionnant et en classant les contenus, en en déterminant la présentation et en augmentant la visibilité de certains d'entre eux au détriment d'autres, les plateformes, par le biais des algorithmes, jouent bien un rôle actif. J'appelle donc une nouvelle fois à une véritable réforme du régime européen de responsabilité des hébergeurs, afin de prendre en compte ce paramètre. Je rappelle d'ailleurs que le Sénat l'avait appelé de ses voeux dans sa résolution

primordial que l'Europe légifère la première, selon ses valeurs et ses principes, pour fixer un « étalon-or » mondial, selon l'expression de France Haugen devant le Parlement européen. Ainsi, nous serons capables d'inspirer d'autres pays. Même si les trilogues qui devraient être lancés en janvier s'annoncent

qui, au dire des industriels français qui y participaient, est aujourd'hui gangréné de l'intérieur par les Gafam ? En effet, la participation des géants américains et, maintenant, de Huawei,

pour garantir notre souveraineté collective et une autonomie stratégique réelle, particulièrement dans les domaines clefs qui vont contribuer à la prospérité de nos peuples ? Mes

nous devons nous interroger sur les limites et les insuffisances des États membres et de l'Union européenne dans le domaine de la santé. Où en est la relocalisation promise de la production de médicaments stratégiques ? Où en est la recherche européenne, notamment pour ce qui concerne les vaccins, dans

tous les États membres et l'Union européenne sont en retard sur leurs principaux concurrents nord-américains, chinois, mais également israéliens et indiens. J'ai déjà eu l'occasion de le souligner, la question de la mise en oeuvre d'un français ou européen est emblématique.

Les objectifs inscrits dans le volet énergie du paquet climat sont particulièrement exigeants pour les États membres, quels que soient les efforts déjà accomplis pour réaliser la transition énergétique. Qu'on en juge : cette transition énergétique suppose de multiplier par deux la production d'électricité à l'échelle du continent ; c'est le défi industriel des prochaines décennies. Or la flambée des prix des énergies démontre aujourd'hui la nécessité de sortir de notre dépendance par rapport aux énergies fossiles et importées. C'est une urgence, dans le domaine tant climatique qu'économique. Il s'agit aussi d'une exigence pour notre transition et notre souveraineté énergétiques. Cette flambée révèle les limites du marché européen de l'énergie. L'indexation des prix de marché de l'électricité sur ceux du gaz, l'extinction des tarifs réglementés pour le gaz ou l'introduction des contrats dynamiques pour l'électricité, prévues par le droit européen, ont d'importantes répercussions pour les consommateurs. Nous attendons du Gouvernement qu'il promeuve une véritable régulation à l'échelon européen, au-delà des déclarations d'intention. Cette flambée révèle aussi les divergences entre États membres. Contrairement à l'Espagne ou à l'Allemagne, la France n'a pas fait le choix d'une baisse massive de la fiscalité énergétique,

Au-delà de cette conjoncture, l'Union européenne doit favoriser les énergies décarbonées sur son territoire. Pour ce faire, elle doit respecter la souveraineté des États membres, seuls compétents pour choisir leur bouquet énergétique selon le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. librement et résolument, définir leurs stratégies industrielles et mobiliser les investissements nécessaires. À cet égard, l'inclusion de l'énergie nucléaire dans la taxonomie européenne sur les investissements durables est absolument cruciale. À l'heure où la France et bien d'autres pays européens font part de leurs intentions d'investir dans le nucléaire, il est impératif de garantir à cette énergie une neutralité technologique, car elle permet de produire une électricité stable, compétitive et peu émettrice de carbone, avec un strict contrôle de la sûreté des installations et de la gestion des déchets. Pour garantir cette neutralité, la production d'électricité nucléaire doit être assimilée non pas à une activité transitoire, voire habilitante, comme pourrait l'être le gaz naturel, mais bien à une activité durable, comme toutes les autres sources d'énergie décarbonée. Convaincu de cette nécessité, le Sénat, sur l'initiative des commissions des affaires économiques et des affaires européennes, vient d'adopter une résolution en ce sens. Nous croyons qu'il est fondamental d'intégrer l'énergie

Il est tout aussi crucial que la taxonomie évite toute distorsion de concurrence entre l'hydrogène nucléaire et l'hydrogène issue des énergies renouvelables. Enfin, la question du calendrier est importante. Nous souhaitons que l'acte délégué attendu soit pris avant la fin de l'année, de sorte qu'il entre en vigueur en même temps que les autres dispositions de la taxonomie. Ce sont ces lignes rouges, fixées par le Sénat dans sa résolution, que nous vous proposons de faire vôtres, monsieur le secrétaire

Cette décision aurait des effets économiques immédiats et une incidence sur les choix énergétiques des États membres. Elle rétablirait un certain équilibre au sein du couple franco-allemand, qui diverge aujourd'hui

nouveaux réacteurs, qui s'élèverait à au moins 46 milliards d'euros selon EDF, les conditions de financement de l'énergie nucléaire auront un impact sur la compétitivité et le coût de la production d'électricité française. En répondant à la flambée des prix et en enrichissant la taxonomie, notre production

L'objectif est de mieux donner aux Européens de tous horizons la possibilité de s'exprimer, afin que leurs attentes influent sur la direction et l'élaboration des futures politiques de l'Union En théorie ... parce que la réalité est tout autre ! Pour grand nombre de nos compatriotes, c'est une Arlésienne ; et pour cause : aucune promotion de cette conférence n'est faite auprès d'eux. Pourtant, les espaces publicitaires ne manquent pas. Nous ne pouvons allumer la radio ou la télévision sans entendre ou voir une campagne publicitaire du Gouvernement faisant la promotion du plan de relance ou de l'entrepreneuriat français. Alors, monsieur le secrétaire d'État, pourquoi ne pas avoir encouragé les Français à se saisir de cet espace d'expression, à se prêter à cet exercice de démocratie participative,

Ma seconde question porte sur les conséquences, pour la défense européenne, du contrat de coalition du futur gouvernement allemand. La lecture de ce document nous confirme la vision atlantiste et circonspecte du gouvernement allemand à l'égard du développement de la défense européenne. preuves : la souveraineté stratégique européenne qui n'intègre pas la question de la défense, le privilège donné à la coopération entre armées nationales et non à une armée européenne, la promotion des stratégies de sortie de conflit et des interventions à titre civil, le choix assumé du passage à la majorité qualifiée pour les décisions du Conseil et, enfin, l'intérêt affirmé pour des relations privilégiées avec les États-Unis dans le cadre d'un agenda renforcé. Ce n'est pas une surprise, mais c'est particulièrement décevant, voire extrêmement énervant, notamment après les crises que nous venons de traverser. Nous avons de quoi être très pessimistes, monsieur le secrétaire Que va devenir le système de combat aérien du futur, le fameux SCAF, aujourd'hui au point mort ? N'était-ce pas une erreur de se concentrer sur la relation franco-allemande, d'écarter l'Italie du SCAF et de laisser l'Espagne se tourner vers les F-35 ?

C'est fort dommageable, car les attentes sont fortes. Oui, la défense aurait pu être un beau projet européen

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, les années passent, les problèmes demeurent ! Crise migratoire, tensions dans l'est de l'Europe, inquiétude vis-à-vis de la Chine, suite du Brexit, difficultés dans le secteur de l'énergie : les dossiers s'accumulent pour la présidence française de l'Union qui se déroulera, cela a été dit, dans un double contexte de l'élection présidentielle et législatives en France et sans doute encore, malheureusement, de pandémie. En matière migratoire, personne ne souhaite revivre les terribles années 2015 et 2016. Pourtant, la situation se dégrade sur les frontières orientales de l'Europe l'Italie est également sous pression. Dans la zone Manche-mer du Nord, une hausse des traversées est constatée depuis plusieurs mois et le préfet maritime vient de faire part d'une nouvelle accélération, en novembre, dans un secteur très dangereux. déroulée au large de Calais illustre les risques mortels courus par les migrants. Certaines communes, de la côte normande aux rivages des Hauts-de-France, sont en première ligne et subissent les désagréments d'un contexte qui dure depuis plusieurs années. Le Royaume-Uni conserve son pouvoir d'attraction. Quand cela l'arrange, il s'accommode des migrants, qui fournissent des travailleurs à bas coût. Dans le même temps, il se prémunit se prémunit à sa manière contre les flux migratoires. La France n'est en définitive qu'un filtre ou une zone tampon. Au même moment, les Britanniques traînent opportunément

flotte qui se préparent constituent en fait le financement d'une mise à la casse de l'outil de travail des pêcheurs ; parfois, cela concerne des navires neufs. Monsieur le secrétaire d'État, comment redonner confiance en l'Europe lorsque les citoyens ont le sentiment que celle-ci se fait duper sans réaction appropriée ? Nos voisins anglais, on les aime bien, mais on sait aussi qu'ils sont habiles en négociation et habitués aux rapports de force. Il faut accroître, je crois, la pression sur les questions migratoires et la pêche, car chacun constate qu'ils gagnent du temps et suivent en fait un programme de politique intérieure. Sur le volet migratoire, je note que beaucoup, par bienveillance, ne perçoivent le sujet que du seul point de vue humanitaire. C'est absolument respectable, mais l'aspect sécuritaire et désormais stratégique des questions migratoires ne peut être tenu pour secondaire. Les pays instrumentalisent les migrants, provoquent le chaos aux frontières pour fragiliser les États membres et l'Union européenne. C'est un moyen, parmi d'autres, de la guerre hybride.

Cette situation conduit à saper les efforts d'accueil et d'intégration des États membres. Elle fait le lit du communautarisme, puis du séparatisme et renforce le contrôle desdites communautés depuis l'étranger. En réaction, et c'est malheureux, le populisme et la radicalité gagnent du terrain. Il nous faut, monsieur le secrétaire d'État, briser ce cycle infernal. En matière écologique, l'Union européenne s'est fixé des objectifs ambitieux, notamment celui de parvenir à la neutralité carbone d'ici à 2050.

Or les banques sont déjà prudentes en raison des règles dites de et de l'activisme des organisations non gouvernementales (ONG). Enfin, des fonds d'investissement internationaux commencent aussi à se désengager de ces activités, qu'ils estiment non durables ou non éthiques.

souveraineté énergétique. Mes chers collègues, je veux terminer par un mot sur la Birmanie ; cela nous éloigne un peu des questions européennes, mais c'est tout de même un véritable sujet. L'Union européenne avait condamné le coup d'État militaire et pris plusieurs séries de sanctions contre la junte et ses intérêts, mais la situation ne semble guère s'améliorer. Il existe un risque de normalisation de la junte ou de glissement vers une guerre civile. Devant le Sénat, le ministre du commerce extérieur avait indiqué qu'aucune piste n'était écartée,

Ce télescopage des calendriers ne me semble pertinent ni pour la France ni pour l'Union européenne. Par ailleurs, au printemps 2022 s'achèvera aussi la Conférence sur l'avenir de l'Europe, lancée le 9 mai 2021 par le Président de la République. Cette conférence se présente comme un exercice de démocratie participative, à l'image du grand débat national en France, dont on a vu, d'ailleurs, les limites. Son objectif est de donner aux citoyens des 27 États membres la possibilité d'exprimer ce qu'ils attendent de l'Union européenne. Je dois dire que nous avons très peu entendu parler de cette campagne en France ; cette consultation semble susciter le désintérêt de nos concitoyens, malgré l'implication forte du Sénat et de sa commission des affaires européennes, qui en a fait la publicité, ainsi que du réseau des « maisons de l'Europe », notamment de celle du département élu. Il est infiniment louable de vouloir recréer du lien entre les institutions et les citoyens européens, mais la confiance dans les institutions démocratiques ne peut être regagnée uniquement par des consultations.

Les institutions européennes, les parlements nationaux et les gouvernements ont la responsabilité de préserver l'ordre européen, afin que l'Europe soit véritablement un espace de liberté, de mobilité, de sécurité, de justice et de solidarité.

La présidence française compte effectivement sur les résultats de cette consultation, ainsi que sur les débats citoyens organisés à l'échelon régional, pour éclairer ses priorités politiques.

plus de droits sociaux en Europe -, la question des valeurs- protéger le droit des femmes, le droit à l'avortement, la liberté de la presse ou encore l'indépendance de la justice -et la puissance de l'Europe. Vous savez combien la question des valeurs est sensible et importante. L'Union européenne vit aujourd'hui un moment critique, mais la crise de la covid-19 l'a renforcée ; je pense par exemple à la gestion mutualisée du vaccin ou à la reprise économique rendue possible grâce au soutien du plan de relance européen. Parallèlement, une prise de conscience a eu lieu et les initiatives se multiplient pour réindustrialiser, relocaliser, accélérer la transition écologique, décarboner notre économie, réduire notre dépendance

Je suis européen et je crois en l'Europe des projets, mais on voit bien qu'il existe une fracture culturelle, avec, à l'ouest, un libéralisme décomplexé et, à l'est, un conservatisme qui s'oppose chaque fois plus au progressisme des sociétés occidentales et qui se braque dès que les institutions communautaires souhaitent inscrire, par exemple, l'avortement ou la non-discrimination sexuelle au rang des « droits inviolables » ou de la « protection des minorités le secrétaire d'État, puisque vous avez affirmé souhaiter que le droit à l'avortement soit intégré à notre socle de droits fondamentaux. Pouvez-vous nous le confirmer ? La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne a été proclamée lors du Conseil européen de Nice, le 7 décembre 2000. Elle comporte 54 articles consacrant les droits fondamentaux des personnes au sein de l'Union européenne, articles qui sont répartis entre les six valeurs constituant le socle de la construction européenne dignité, liberté, égalité, solidarité, citoyenneté et justice. L'Union européenne est unie dans la diversité, mais il semble indispensable que l'Europe réaffirme les valeurs qui fondent sa civilisation face au reste du monde. Le Gouvernement s'est fortement impliqué sur la question du respect des droits dans certains pays de l'Union européenne. Veuillez

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, la prochaine réunion du Conseil européen fera le point sur les travaux visant à renforcer notre préparation, notre capacité de réaction ainsi que notre résilience collective face aux crises à venir, et à protéger le fonctionnement du marché intérieur. La réponse apportée par l'Union européenne à la pandémie a démontré sa valeur ajoutée, par exemple avec les résultats positifs concernant la production, l'acquisition et la répartition des vaccins. Toutefois, la pandémie a aussi mis en lumière les défaillances de l'Union européenne sur le plan de la préparation et de la réaction aux crises multisectorielles. L'union est encore insuffisamment prête pour faire face à des crises graves de nature différente, qui pourraient être multidimensionnelles, hybrides, avoir des effets en cascade ou se produire simultanément. En 2013, le Conseil européen a créé un dispositif intégré pour une réaction au niveau politique dans les situations de crise, dit IPCR, qui a récemment été activé dans le cadre de la crise migratoire et de la crise sanitaire.

mais, incontestablement, il faut mettre en oeuvre la mise à jour de la stratégie industrielle de l'Union européenne présentée en mai dernier, notamment pour diversifier les chaînes d'approvisionnement et forger de nouvelles alliances industrielles. Cela permettra de réduire la dépendance de l'Union à l'égard de certains pays tiers, notamment dans les secteurs jugés critiques : matières premières, substances actives pharmaceutiques ou encore produits essentiels pour soutenir la double transition verte et numérique comme les semi-conducteurs. Depuis plusieurs mois, partout dans le monde, les entreprises sont confrontées à des pénuries de matières premières et de produits semi-finis ; métaux, bois, papier, aluminium, plastique, blé ou encore semi-conducteurs : la liste s'allonge au fil des semaines. couplées à l'augmentation des prix de l'énergie, freinent la reprise de l'activité industrielle, alimentent l'inflation et pèsent sur les budgets des ménages. La pandémie a mis en lumière nos fragilités. Une réflexion essentielle s'est engagée sur la question de la relocalisation de certaines productions et sur l'accès de l'Europe aux ressources. La Commission européenne a notamment présenté, voilà un an, un plan d'action sur les matières premières critiques pour les secteurs stratégiques et lancé de nouvelles alliances industrielles.

La pénurie actuelle de semi-conducteurs a par ailleurs mis en évidence le rôle fondamental de ces composants, indispensables pour tous les secteurs- ils sont toujours plus nombreux -qui utilisent des équipements électroniques. Ainsi, le président américain annonçait en avril dernier un plan de 50 milliards de dollars pour soutenir et développer ce secteur stratégique. En juillet, la Commission lui répondait en lançant une alliance industrielle pour les processeurs et les semi-conducteurs, afin que l'Europe atteigne au moins 20 % de la production mondiale.

Monsieur le secrétaire d'État, pouvez-vous nous préciser les contours de cette future législation et, surtout, nous éclairer sur sa complémentarité avec l'alliance industrielle, qui commence à peine à se structurer ? Par ailleurs, le Conseil européen reviendra sur les évolutions récentes concernant les prix de l'énergie. Je veux m'y arrêter un instant pour finir. la Commission européenne a présenté une « boîte à outils » visant à aider les États membres à atténuer l'impact de la flambée des prix de l'énergie sur les ménages et les entreprises, ne prévoyant pas de nouvelle initiative européenne particulière. Elle n'a pas donné suite à la demande de la France de réviser le fonctionnement du marché européen de l'électricité, qui aboutit de fait à arrimer le prix de l'électricité à celui du gaz. Or la France, qui dispose de nombreuses centrales nucléaires, souhaite découpler le prix de l'électricité de celui du gaz, ce qui lui permettrait de proposer une électricité encore moins chère, mais neuf États membres s'opposent fermement à cette demande et soutiennent les « principes concurrentiels de la conception de nos marchés de l'électricité et du gaz », jugeant la hausse des prix seulement conjoncturelle. Aux côtés de l'Espagne, de l'Italie, de la Grèce et de la Roumanie, la France réclame une modification de la directive sur le marché intérieur de l'électricité, afin notamment de permettre aux États membres d'appliquer des mécanismes de régulation garantissant que les prix de l'électricité reflètent les coûts du mix de production utilisé par le pays.

équilibrée, renforcée en matière policière et judiciaire avec le Royaume-Uni. Un cadre européen et un cadre large : telles sont les deux conditions que nous avons toujours posées. En effet, et je termine ma réponse

irréversibles. Nous aurons des moments de doute, nous aurons des moments d'inquiétude sur le plan industriel, mais il faut saluer ce choix stratégique qu'ont fait en 2017 la chancelière Merkel et le président Macron, après le Brexit. On ne peut pas construire une politique de sécurité et de défense européenne sans se lancer dans des projets industriels communs qui formeront l'ossature

pleinement cette présidence française de l'Union européenne. Pour la première fois, je tiens à le souligner, j'ai réuni à quatre reprises- et je continuerai de le faire -un comité transpartisan composé d'un représentant de chacun des groupes politiques de

pour faire durablement adhérer nos concitoyens au projet européen. Si ce projet n'est qu'un projet de marché, qu'un projet de budget, il ne suscitera pas d'adhésion politique, quoi qu'on pense de l'Europe, avec des sensibilités qui peuvent être très différentes. Dans tout